j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Gérard Claudel, qui fut sénateur du Val-d'Oise de mai à septembre 2004.

donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe

de la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. J'ai déjà insisté dans cet hémicycle, voilà quelques semaines, sur l'utilité de ce texte. ce texte. Nos concitoyens guadeloupéens connaissent d'inacceptables difficultés dans leur accès à une ressource aussi essentielle que l'eau potable. Il nous fallait donc agir avec célérité et efficacité : c'est l'ambition de cette proposition de loi. Le texte retenu par la commission mixte paritaire est, pour l'essentiel, sous réserve de rares modifications rédactionnelles, celui qu'a élaboré et voté le Sénat lors de sa séance du 10 mars dernier. Cette proposition de loi, déposée, en des termes similaires, par la députée Justine Benin et notre collègue Dominique Théophile, a donc été utilement enrichie et complétée lors de son examen par notre assemblée. Je m'en félicite. Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, la proposition de loi posait d'ores et déjà le principe d'un syndicat mixte unique de gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement de Guadeloupe et en prévoyait les principales modalités de fonctionnement. Les débats de l'Assemblée nationale avaient surtout été l'occasion de garantir la pleine association des usagers de ces services en prévoyant la création d'une commission de surveillance, chargée d'émettre des avis sur l'exercice par le syndicat mixte unique de ses compétences. L'examen par notre assemblée a été l'occasion, outre l'apport de modifications de nature rédactionnelle, de parfaire le fonctionnement de ce syndicat mixte unique. outre, il nous a semblé nécessaire de permettre à de nouveaux membres de rejoindre, s'ils le souhaitent, le syndicat mixte unique ainsi créé. Encadrée par l'autorisation du préfet et l'accord unanime des membres, cette procédure permettra d'éviter, dans l'éventualité où un tel cas se présenterait, une nouvelle modification législative. ailleurs, nous avons prévu de permettre au comité syndical de décider, à l'unanimité des membres, de déroger à la clé de répartition des contributions financières afin de prémunir le syndicat mixte d'une rigidité excessive dans ses décisions dans ses décisions d'investissement. L'examen du texte au Sénat a également été l'occasion de renforcer les attributions de la commission de surveillance, prévue à l'article 2 de la proposition de loi, et d'en modifier la composition. Le texte issu de la commission mixte paritaire conserve, en la matière, deux apports significatifs du Sénat ainsi, nous avons souhaité assurer une meilleure représentation des élus municipaux au sein de la commission de surveillance et permettre à des personnalités qualifiées d'y siéger. Dans le même esprit, nous avons prévu l'obligation d'une audition annuelle du président du comité syndical par la commission de surveillance. Ces dispositions sont essentielles afin de restaurer la confiance des usagers, majoritaires au sein de la commission de surveillance, dans les services publics de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Ainsi enrichie, la proposition de loi a recueilli le plein assentiment de nos collègues députés. Je souhaite ainsi les remercier pour l'esprit de consensus et d'efficacité dans lequel ils ont inscrit les travaux de notre commission mixte paritaire. Je salue tout particulièrement Justine Benin, signataire et rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, pour nos échanges constructifs. Je remercie également notre collègue Dominique Théophile pour son travail de sensibilisation, au sein de notre assemblée comme en dehors de cette enceinte, sur cette question. Le texte adopté par la commission mixte paritaire apportant une réponse rapide et pragmatique à un problème qui n'a que trop duré, je vous invite, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire. La satisfaction d'un travail législatif consensuel et de qualité n'équivaudra néanmoins pas à donner quitus au Gouvernement sur cette question. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, j'ai eu l'occasion de rappeler que ce texte, bien qu'utilement enrichi, ne constituera qu'un premier pas dans la résolution d'une situation particulièrement complexe. Nous sommes parfaitement conscients qu'il ne suffira pas, à lui seul, ni à restaurer la confiance des Guadeloupéens dans leurs services publics ni à résoudre les problèmes qu'ils déplorent au quotidien. L'amélioration de l'accès à l'eau pour nos concitoyens guadeloupéens suppose en effet de mettre en oeuvre d'autres mesures, qui ne relèvent pas du domaine législatif. Le législateur a fait sa part ; il revient désormais à l'ensemble des acteurs de se saisir des outils ainsi mis à leur disposition. Je me tourne vers vous, monsieur le ministre : l'État doit se montrer à la hauteur du mécontentement des Guadeloupéens et des attentes générées par cette proposition de loi. Ce texte ne dispensera pas le Gouvernement, qui dispose des moyens humains, techniques et financiers de l'État, d'agir rapidement et efficacement pour nos compatriotes guadeloupéens. Notre assemblée sera vigilante, monsieur le ministre, à ce que ce souhait, que je formule devant vous solennellement, ne demeure pas un voeu pieux. Très bien

les problèmes d'organisation d'une compétence- le ministre Lurel et le sénateur Théophile savent que je dis cela avec beaucoup de respect et de prudence, car il faut défendre les élus locaux et la démocratie représentative.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous ici : depuis plusieurs années, la gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens guadeloupéens. Ce sont ainsi près de 100 000 usagers qui sont régulièrement victimes de « tours d'eau », suscitant colère et exaspération. Cette situation est d'autant plus difficile à accepter qu'elle ne résulte pas de causes naturelles propres à la Guadeloupe, où la ressource en eau est abondante. Un des principaux problèmes réside dans le caractère éclaté de la gestion des services d'eau et d'assainissement, qui fait obstacle à la gouvernance d'ensemble dont la Guadeloupe a besoin. En outre, les syndicats compétents sont dans une situation difficile la plupart d'entre eux ne peuvent ni effectuer les investissements nécessaires à l'entretien et à l'amélioration du réseau, ni entreprendre les travaux d'urgence, ni payer les fournisseurs. Il apparaît donc crucial et urgent d'unifier la gouvernance de la gestion des services publics d'eau et d'assainissement en Guadeloupe, car nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes souffrir davantage d'une telle indignité. Aussi, cette proposition de loi, qui a été discutée et enrichie par nos deux assemblées, concourt à répondre à une situation inacceptable et persistante. C'est pourquoi je me réjouis que la commission mixte paritaire se soit déroulée dans un esprit de recherche de complémentarité et de consensus et qu'elle ait abouti à un texte commun. Je me félicite également que le Sénat ait apporté de nombreuses modifications afin d'améliorer l'effectivité des dispositions de cette proposition de loi. Le Sénat a ainsi enrichi l'article 1 d'un certain nombre d'assouplissements. Je veux parler de la possibilité pour une autre personne publique d'adhérer au syndicat mixte, après accord unanime de ses membres et accord exprès du représentant de l'État en Guadeloupe. Je veux également évoquer la possibilité pour le comité syndical de déroger, après accord unanime de ses membres, à la répartition des contributions financières lorsqu'un projet d'investissement le nécessite. Je veux enfin mentionner la possibilité, pour le syndicat mixte, d'étudier la faisabilité d'une tarification sociale de l'eau. Concernant l'article 2, qui prévoit la constitution d'une commission de surveillance auprès du syndicat mixte, le Sénat a souhaité rationaliser la composition de celle-ci, notamment en prévoyant la présence de représentants des communes et de personnalités qualifiées et en supprimant la présence des parlementaires en son sein. Il a, par ailleurs, prévu une audition annuelle et obligatoire du président du comité syndical par la commission de surveillance, de façon à favoriser la fluidité entre leurs travaux. Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de notre collègue Françoise Dumont, qui a oeuvré de façon constructive pour élaborer un texte commun si important pour la Guadeloupe. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi constitue une étape importante vers la résolution d'une situation complexe et inacceptable pour les Guadeloupéens. et Territoires votera ce texte, lequel apportera une première réponse concrète et pragmatique aux multiples dysfonctionnements auxquels sont confrontés les services publics de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous partageons le constat : la situation de l'eau en Guadeloupe est un problème à bien des égards- citoyens sujets à de nombreuses coupures, dépenses trop importantes, gaspillage de la ressource, non-entretien du réseau, dette abyssale des structures gestionnaires, tarification et facturation opaques. Il était plus qu'urgent d'agir au bénéfice des usagers, d'agir contre le gaspillage de l'eau et d'améliorer véritablement la qualité de celle-ci. Si plusieurs initiatives se sont succédé afin de résoudre ces difficultés, rien n'avait permis, à ce jour, d'envisager une réelle restructuration pérenne, apte à résoudre les problèmes structurels du système de gestion de l'eau en Guadeloupe.

concrète que permet ce texte est certes nécessaire, mais pas suffisante : il est urgent de réagir et de permettre un moindre gaspillage de l'eau pour les usagers, tout comme une amélioration forte de sa qualité.

le volume d'eau consommé était de 26,4 millions de m, alors que 73,1 millions de m étaient produits. » Les pertes représentent donc 177 % de la consommation. Ses conclusions sont sans appel : pour un litre d'eau consommé, un litre et demi de perdu, ce qui entraîne une pression bien trop importante sur les ressources comme les eaux souterraines du Nord Grande-Terre. De plus, la qualité de l'eau est « inquiétante », en raison « du très mauvais niveau d'assainissement et de l'utilisation historique de polluants » comme le chlordécone. Pour la Guadeloupe, le GREC a aussi mis en avant de possibles problèmes de sécheresse en se fondant sur des prévisions de précipitations qui diminueront dans une large partie des zones habitées. large partie des zones habitées. L'article 1 met en place une autorité unique, sous une forme proche d'un syndicat mixte dirigé par un comité syndical. Il conserve deux apports sénatoriaux majeurs.

Cette réforme ne sera que le premier pas important d'une gestion durable de l'eau en Guadeloupe. En ce qui concerne le financement et les modalités de transition entre les deux systèmes, notre groupe reste prudent et attend un engagement financier fort de l'État, comme nous l'avons rappelé en première lecture. Notre groupe appelle à la plus grande vigilance sur le transfert des dettes actuelles à la nouvelle structure. Une attention particulière devra être portée au volume des dettes transférées, ainsi qu'aux dettes qui resteraient à la charge des entités actuelles.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la commission mixte paritaire réunie le 23 mars dernier est donc parvenue à un accord sur la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Les quelques dispositions qui restaient en discussion ont fait l'objet d'un consensus que nous saluons et qui reflète l'esprit dans lequel la députée Justine Benin et moi-même avons souhaité inscrire ces débats. Nous avons eu l'occasion, ces dernières semaines, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, de décrire les dysfonctionnements qui ont entaché nos services publics, ainsi que leurs conséquences sur notre économie, sur notre système de santé ou sur notre environnement. Il n'est plus utile d'y revenir. La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui- vraisemblablement pour la dernière fois -entend satisfaire une revendication ancienne, portée par les élus locaux et les forces vives de notre territoire, à savoir la création d'une structure unique consacrée à la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Plusieurs rapports et audits, dont celui du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), en mai 2018, ont d'ailleurs démontré la pertinence de ce projet. Ce texte est le fruit d'un travail collectif qu'il convient de rappeler brièvement. Il se veut d'abord fidèle aux échanges et aux attentes des élus, des associations d'usagers et des Guadeloupéens, que nous avons rencontrés régulièrement, et des semaines durant, avec ma collègue Justine Benin. À l'Assemblée nationale, les députés ont enregistré un certain nombre d'avancées. C'est le cas de la création d'une commission de surveillance, en lieu et place de la commission consultative initialement envisagée, afin de garantir la juste représentation des usagers et de tenter de retrouver une confiance aujourd'hui perdue. C'est le cas également du compromis trouvé avec le Gouvernement sur la question des dettes fournisseurs. Au Sénat, le travail de Mme la rapporteure Françoise Dumont et de l'ensemble de nos collègues a permis d'apporter, pour ne citer que ces quelques exemples, davantage de souplesse au fonctionnement du comité syndical et de renforcer les prérogatives de la commission de surveillance. Ces apports dans leur grande majorité par la commission mixte paritaire, preuve, s'il en fallait une, de la qualité des échanges et des travaux menés par nos deux assemblées. Si le texte qui nous revient aujourd'hui et sur lequel nous nous prononcerons dans quelques instants est un préalable à la remise en état du système de distribution d'eau potable en Guadeloupe, il n'en demeure pas moins une étape. Cette étape ne pourra seule résoudre les difficultés que nous connaissons. Plusieurs chantiers s'ouvriront donc dans les jours et les semaines qui viennent. Il s'agira de clarifier le traitement de la ressource pour assurer une gestion durable de notre sous-sol, de mobiliser des financements pour assurer à ce syndicat un fonctionnement pérenne et, enfin, de définir et de réaliser les investissements les plus urgents. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des élus guadeloupéens, qu'ils soient municipaux, communautaires, départementaux ou régionaux, les syndicats et les associations d'usagers, ainsi que le personnel affecté aux services d'eau potable et d'assainissement, que je sais motivé et qui doit trouver toute sa place dans cette nouvelle structure, à créer dès à présent les conditions de sa mise en oeuvre. Le chantier qui s'annonce est immense, mais il est nécessaire et ô combien salutaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, chacun d'entre nous avait pu faire état, déjà lors de la première lecture, de son inquiétude, voire de sa stupéfaction, face aux différents rapports, bilans et analyses sur la situation du service public de l'eau potable en Guadeloupe. Je n'y reviendrai pas dans le détail. Toutefois, je veux redire, comme l'avait fait notre collègue président de la délégation aux outre-mer, Stéphane Artano, combien il est inacceptable que, en 2021, certains de nos concitoyens aient des difficultés d'accès à l'eau potable, non pas en raison d'une catastrophe soudaine, mais à cause d'un réseau en mauvais état et d'une gestion désastreuse. La France de l'outre-mer ne saurait être une oubliée de la République. Face à cela, le principe de la libre administration des collectivités territoriales doit donc céder. En effet, pour qu'il puisse être pleinement efficace, il faut qu'en cas de défaillance l'État reprenne la main. Pourvu, cependant, que ce recours à la loi demeure occasionnel ! Ce sera à nous d'y veiller. Tel est l'objet de cette proposition de loi : apporter un correctif à un service que la liberté locale n'a pas pu ou su faire fonctionner. Cependant, il est plus que regrettable que cela ait touché durant plusieurs années un service aussi essentiel que celui de la gestion de l'eau potable. En réponse à une telle situation, le consensus de nos deux assemblées dans le cadre de la commission mixte paritaire est une première satisfaction. Le sujet était trop important pour que nous ne puissions pas y parvenir. Nous répondrons dans l'unité aux Guadeloupéens qui subissent cette situation. Aussi, les solutions proposées sont satisfaisantes, en permettant la création d'un syndicat mixte et d'une commission de surveillance. Ces deux institutions laissent espérer, tant à court qu'à long terme, une restauration du service public au travers d'une mutualisation et d'une unification de sa gouvernance. Du point de vue du syndicat mixte, nous pouvons nous réjouir que certaines souplesses aient été introduites au cours de la navette parlementaire. Si la loi doit intervenir pour pallier les carences de la libre administration locale, elle doit le faire avec mesure, notamment en permettant à de nouveaux membres de bénéficier à l'avenir des apports de ce nouveau système. S'agissant, ensuite, de la commission de surveillance, elle permettra d'associer l'ensemble des acteurs locaux dans la gestion du service. Le Sénat avait proposé certains ajustements concernant sa composition ; ils ont été retenus dans ce texte. Je pense notamment au retrait des parlementaires. En effet, chacun doit demeurer dans ses fonctions et cette présence n'était pas nécessairement judicieuse, d'autant que,

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas encore nous féliciter du travail accompli, dans la mesure où il ne s'agit que d'une première étape dans un processus long et laborieux. Ces seules institutions ne suffiront pas à régler toutes les difficultés de l'accès à l'eau potable en Guadeloupe. Le groupe RDSE votera donc en faveur de ce texte, mais fera preuve d'une vigilance particulièrement accrue au cours de ces prochaines années, afin de veiller à ce que ce territoire de la République ne demeure pas enlisé dans cette crise. La parole

Varaillas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte arrêté en commission mixte paritaire permet de conserver des apports du Sénat, afin de rendre un peu plus souple le fonctionnement du syndicat mixte créé par la présente proposition de loi ou encore d'intégrer une réflexion sur la tarification sociale de l'eau, qui est un impératif de justice sociale. Toutefois, nous estimons que cette structure imposée d'en haut aux Guadeloupéens demeure très contraignante et l'obligation pour l'ensemble des communautés d'agglomération d'y adhérer en est emblématique. Une telle dépossession des compétences des EPCI peut être interprétée comme une ingérence importante de l'État dans la libre administration des collectivités, surtout dans un contexte local de négociation entre les acteurs intéressés. Une « feuille de route » a été adressée aux élus locaux par le Gouvernement. Elle est vécue par beaucoup comme une mise sous tutelle et une mise à l'écart de l'expertise guadeloupéenne. La crainte du retour des multinationales pour gérer la production et la distribution de l'eau et la nécessité de recueillir une aide financière renforcent la pression sur les élus. Ce consensus forcé pour aboutir à une entité formelle ne garantit en rien son bon fonctionnement et la manière dont le syndicat s'intégrera au préexistant. Nous le répétons, la forme est là, mais le fond nous questionne. En effet, plusieurs interrogations demeurent. S'agissant du financement du département et de la région, l'État s'est engagé à ne pas alourdir le budget des collectivités du fait de dépenses nouvelles. Mais comment compte-t-il concrétiser cet engagement ? Les élus locaux ne peuvent se contenter de promesses tant ils savent par ailleurs l'érosion dans le temps des compensations financières de l'État. Les principales dettes des EPCI devront être transférées au nouveau syndicat pour éviter que cette instance soit mort-née. La question est toujours latente et les élus attendent des réponses. L'avenir des salariés des structures actuelles n'est toujours pas clair. Des garanties devront être apportées, pour que chacun puisse retrouver un emploi au sein de la nouvelle structure. Sur le terrain, le comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe ne se satisfait pas du texte. Il a récemment demandé un référendum sur le sujet et souhaite que les usagers soient mieux impliqués dans le processus de gouvernance de l'eau. Ses réclamations portent sur le montant excessif des factures envoyées aux usagers, l'instauration d'un tarif équitable pour tous et l'arrêt des poursuites judiciaires, alors que les services sont défaillants. Le sujet en toile de fond de ce texte est celui de l'accès à l'eau et de la raréfaction des ressources en eau, qui touche en premier les territoires marins et nécessite l'appel à la solidarité nationale et internationale. Les collectivités d'outre-mer sont impactées par des réseaux vétustes, où plus de la moitié de l'eau se perd dans les fuites. Pourtant, les habitants, dont le quotidien est rythmé par des coupures d'eau, continuent de payer des factures. L'eau est un bien commun essentiel à la vie impliquant des enjeux écologiques, sociaux et économiques, d'où l'importance d'une gestion publique pour garantir son accès, mais également sa qualité. Alors que le droit à l'eau et à un assainissement de qualité a été reconnu par l'ONU en 2010 comme « un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme », ce droit est bafoué et les inégalités liées à cette ressource s'aggravent. Le 15 avril prochain, notre groupe proposera de faire de ce droit à l'eau, aujourd'hui fictif, un droit réel. Nous défendrons, dans le cadre d'une proposition de loi, un accès pour toutes et tous à l'eau potable et à l'assainissement. Nous défendrons la gratuité des premiers litres d'eau nécessaires au quotidien, nécessaires à la vie. Présentement, nous restons dubitatifs, il faut bien le dire, pour ce qui concerne le schéma proposé pour la gouvernance du service d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, sur les plans tant administratif que financier. Nous maintenons donc notre position d'abstention sur ce texte.

Le fait que la question des ressources humaines ne soit pas traitée constitue pour nous un élément de surprise. Nous y voyons des difficultés à venir. Nous

Monsieur le ministre, vous portez ce texte avec beaucoup d'ambition et dynamisme. Je le rappelle, le « quoi qu'il en coûte » concerne le traitement de la pandémie ; il ne semble pas avoir vocation

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je l'avoue, en venant à cette tribune, je suis un peu partagé.

ancien ministre de l'outre-mer, a dit tout l'attachement qu'il portait à l'actuel ministre de l'outre-mer, qu'il me soit permis de dire tout le bien que je pense de notre rapporteure pour tout le travail qu'elle a accompli. Tout le monde ici aura compris la nécessité

Victorin Lurel, l'inclusion de l'évaluation des possibilités d'une tarification sociale, dont vous vous êtes fait écho ici même avec notre collègue Victoire Jasmin.

Je partage les inquiétudes exprimées par notre collègue Philippe Bonnecarrère, car je me méfie toujours des structures qui épousent tout ce que nos institutions comptent de collectivités. En effet, à un moment donné, il faut prendre des décisions.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.

Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, mesdames, messieurs les sénateurs, le sujet de la formation des élus locaux, qui nous rassemble aujourd'hui, constitue un enjeu essentiel au bon fonctionnement de notre vie démocratique. Ce sujet me tient particulièrement à coeur

et moi-même, qui a créé notamment le droit individuel à la formation des élus locaux. Nous savons tous ici ce que la fonction d'élu local suppose d'exigences,

de leur permettre d'être mieux « armés » dans l'exercice de leur fonction d'élu, ce qui appelle une formation bien différente d'une formation professionnelle classique. Deux principes doivent être garantis : la pluralité de l'offre-

habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet. Après avoir rendu public un rapport d'inspection aux constats parfois préoccupants, nous avons lancé un vaste cycle de concertations, avec, d'une part, les associations nationales d'élus, et, d'autre part, les organismes de formation agréés. Je veux ici les remercier de leur implication. Cette concertation a conduit à un projet d'ordonnance sur lequel le Conseil national d'évaluation des normes a rendu un avis favorable unanime. Ce n'est pas si fréquent ! Permettez-moi de revenir en quelques mots sur les caractéristiques du système actuel et sur ses limites, qui sont l'objet de cette réforme. Tout d'abord, les organismes de formation doivent disposer d'un agrément ministériel pour former des élus. Cet agrément n'a, hélas, pas permis d'éviter des dérives dans le secteur. Ensuite, la formation des élus est financée par deux dispositifs complémentaires. Depuis 1992, les collectivités doivent prévoir un budget de formation de leurs élus, égal au minimum à 2 % des indemnités qui peuvent leur être versées. Ce budget minimum devrait représenter au moins 34 millions d'euros. Mais les petites communes n'ont parfois pas les moyens nécessaires pour faire face aux demandes.

Ils disposent, à ce titre, de vingt heures de formation par an cumulables. Ce droit est financé par une cotisation d'un montant égal à 1 % des indemnités versées aux élus, ce qui représente environ 16 millions d'euros. Force est de constater un certain nombre de dérives par rapport à l'esprit de la loi : prix élevés, faible nombre d'élus formés, concentration de la dépense sur quelques organismes, déficit très important. La réforme dont nous allons discuter s'attaque à chacun de ces sujets. Premièrement, l'ordonnance conforte le dispositif de financement par les collectivités, auquel celles-ci sont très attachées. Pour répondre Pour répondre aux besoins des petites communes, l'intercommunalité à fiscalité propre pourra désormais, selon des modalités absolument souples, contribuer à la formation des conseillers municipaux, sans exercer cette compétence En outre, une collectivité pourra désormais abonder très facilement le compte DIFE de l'élu, afin qu'il puisse cumuler aisément les deux sources de financement.

je pèse mes mots -à présenter leur offre de formation comme « gratuite », alors qu'elle coûtait en réalité de plus en plus en cher. Oui ! L'ordonnance prévoit donc de doter annuellement chaque élu d'une enveloppe en euros. L'élu pourra ainsi choisir le meilleur rapport qualité-prix et se former deux fois plus longtemps s'il choisit un organisme de formation deux fois moins cher. Il aura accès à une vision d'ensemble de l'offre grâce à l'intégration du DIFE dans la plateforme « moncompteformation.gouv.fr », qui gère déjà le compte personnel de formation. La procédure d'inscription sera accélérée. Les frais de gestion seront réduits. Ce dispositif continuera de reposer sur la Caisse des dépôts et consignations, dont je veux saluer l'engagement dans cette réforme. est des formations de réinsertion professionnelle, l'élu pourra facilement cumuler les droits acquis dans le cadre de sa vie professionnelle, de ses engagements bénévoles et de son mandat d'élu, ainsi que les différents compléments de financement qui existent en matière de formation professionnelle de droit commun. Cette réforme est aussi, tout simplement, une opération de sauvetage du DIFE,

À moyen terme, l'équilibre financier sera garanti par la faculté donnée au pouvoir réglementaire, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, de modifier les conditions d'organisation des formations, de moduler le taux de cotisation ou de moduler l'enveloppe accordée annuellement aux élus. Cette enveloppe sera fixée dans la concertation, de manière transparente, en divisant les ressources disponibles par le nombre d'élus demandeurs. Sur ce point, votre rapporteur a déposé, au nom de la commission des lois, deux amendements auxquels le Gouvernement est favorable et dont il partage complètement les objectifs. Le premier vise à garantir la stabilité de l'enveloppe annuelle accordée aux élus pour trois ans, à compter de 2023. Le second a pour objet de prévoir la conversion en euros des heures non utilisées à l'issue de la période transitoire de six mois prévue par l'ordonnance. Ce montant issu de la conversion s'ajouterait à l'enveloppe annuelle en euros qui sera accordée de manière identique à tous les élus locaux. Il convient de garder à l'esprit que les droits en euros du DIFE s'ajouteront aux financements que pourront accorder les collectivités et les intercommunalités, soit en prenant directement en charge une formation soit en abondant le compte DIFE de l'élu. Troisièmement, cette réforme devrait permettre de garantir des formations de qualité, délivrées par des organismes rigoureux. Un répertoire national de la formation des élus sera élaboré de manière concertée, afin de cerner les sujets de formation éligibles au financement public.

Les organismes de formation des élus seront désormais soumis au même statut, et aux mêmes obligations, que les organismes de formation de droit commun. L'ordonnance formalise en outre la procédure de retrait de l'agrément en cas de manquement de l'organisme à ses obligations. ses obligations. Quatrièmement, et enfin, la gouvernance du secteur sera simplifiée et renforcée. L'ordonnance conforte le CNFEL, qui reprendra les missions de la commission DIFE, en lui confiant tous les leviers nécessaires pour rendre des avis parfaitement informés sur l'ensemble des enjeux de la formation des élus. Le CNFEL bénéficiera également des avis d'un conseil d'orientation placé auprès de lui, dans lequel seront notamment représentés les organismes de formation. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, la réforme que le Gouvernement soumet à votre approbation. Mme la rapporteure et la commission des lois, dont je tiens à saluer le travail, ont apporté des amendements utiles au texte du Gouvernement dont elles partagent, me semble-t-il, les objectifs. La discussion qui s'ouvre sur ce texte nous permettra, j'en suis certaine, d'avancer vers une réforme qui confortera la formation des élus locaux. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues,

de sécuriser les choses. Quand vous signez un contrat de formation avec un organisme, vous devez savoir qui va dispenser la formation, et celle-ci ne doit pas être déléguée à un organisme X ou Y qui ne serait pas agréé. Nous proposons

le droit individuel à la formation étant fait essentiellement pour la reconversion, on sait bien que c'est en fin de mandat, au bout de six ans, que les élus consomment les crédits, ce qui provoque une concentration de de la demande. Et nous n'avons pas de visibilité. Il est extrêmement important, pour les organismes de formation, qui sont aussi des employeurs, comme pour les collectivités, de connaître à un horizon de trois ans le montant du crédit en euros dont chaque élu pourra bénéficier.

En effet, parce que le retrait progressif de l'État d'un certain nombre de missions qu'il exerçait dans les territoires s'accentuait, le besoin d'ingénierie territoriale a crû peu à peu. C'est ainsi que nous avons accompagné les 816 maires de l'Aisne,

que vous présidiez à l'époque, madame la ministre, je commettais un rapport intitulé, assorti de la conclusion suivante : « La formation, en ce qu'elle permet une amélioration des connaissances, des compétences et des aptitudes, constitue un outil qui répond à la fois aux intérêts des élus et des agents des collectivités territoriales. En ce sens, le droit à la formation doit être préservé et consolidé. » J'y formulais une quinzaine de propositions, dont bon nombre ont finalement été intégrées dans notre droit, par exemple l'instauration d'un plancher de crédits budgétaires consacrés à la formation, ou encore la mise en place d'un droit individuel à la formation, le DIFE,

rapport intitulé. Complexification du droit, augmentation des compétences des collectivités au fur et à mesure de la décentralisation, montée des intercommunalités : voilà en effet autant de dynamiques qui ont fait de la formation des élus et des agents publics un défi pour l'avenir des collectivités territoriales. C'est donc peu de dire que la formation des élus est un serpent de mer, indissociable de celui du statut de l'élu. Si nous avons pu avancer sur ce dernier point depuis quelque temps, la formation reste un défi majeur et crucial, car la compétence des élus locaux est la véritable condition d'un bon exercice du mandat. Elle permet de compenser les inégalités de formation initiale et elle est devenue une condition de la démocratisation de l'accès aux fonctions politiques. Former les élus, c'est aussi les préparer à l'après-mandat- vous y avez fait référence, madame la ministre. À l'heure où plus personne n'envisage qu'un élu local occupe un mandat toute sa vie, la sortie du mandat et la reconversion supposent une formation adaptée et une bonne préparation en amont.

Cette ratification tardive, bien au-delà des délais impartis, nous aura fait perdre un temps précieux, d'autant que le personnel élu a entre-temps été en partie renouvelé à l'occasion des élections municipales de 2020.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France compte environ 510 000 élus locaux. Pour faire face à leurs lourdes responsabilités et exercer efficacement leurs fonctions, les élus doivent être correctement formés. En outre, il paraît important, pour préserver l'attractivité des fonctions électives, que les élus qui le souhaitent puissent s'inscrire dans un processus de réinsertion professionnelle à la fin de leur mandat. La loi a ainsi prévu deux dispositifs pour répondre aux besoins des élus locaux en matière de formation. Le premier, introduit en 1992, prévoit le financement des formations demandées par les collectivités territoriales, qui doivent inscrire à leur budget chaque année un montant minimum équivalent à 2 % des indemnités dues aux élus. des élus, ou DIFE, introduit en 2015, est financé par un fonds national, alimenté par 1 % des indemnités perçues par les élus indemnisés, soit une somme de 17 millions d'euros annuels. Or ce dispositif n'a pas réussi à garantir des formations de qualité facturées au juste prix ; de nombreux exemples d'abus et de dérives ont été constatés. Le fonds DIFE géré par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, s'est trouvé dans une impasse financière

Vous en conviendrez, il existe une véritable urgence à réformer le dispositif de formation des élus locaux. Dans le cadre de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique,

Le projet de loi qui nous est soumis vise à ratifier deux ordonnances prises sur le fondement de l'article 105 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ces ordonnances visent non seulement à faciliter l'accès à la formation et à garantir la qualité des formations dispensées, mais également à rénover la gouvernance du système de formation des élus locaux. Elles apporteraient ainsi une amélioration certaine et bienvenue. Par ailleurs, je me félicite des travaux en commission, qui ont enrichi le dispositif. De nombreuses dispositions vont dans le bon sens. Je veux parler, tout d'abord, du rétablissement du cumul des droits à la formation des élus locaux sur toute la durée du mandat, afin de leur permettre d'utiliser leurs droits acquis sur plusieurs années, à l'instar du fonctionnement du compte personnel de formation des salariés. Je veux parler également de l'extension des possibilités d'abondements complémentaires par des personnes publiques telles que l'État, Pôle emploi et d'autres collectivités territoriales, afin qu'elles puissent cofinancer les formations à la reconversion des élus locaux déjà financées partiellement par le DIFE. enfin de la possibilité offerte aux élus locaux de s'inscrire, dès la première année de leur mandat et gratuitement, à des modules de formations pouvant être accessibles à distance la plateforme numérique et leur permettant d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de leur mandat. De même, il était particulièrement nécessaire d'approfondir le contrôle des organismes de formation. À cet égard, je me réjouis qu'un certain nombre de dispositions concernant les conditions de sous-traitance par les organismes de formation agréés aient été introduites, afin de garantir la qualité des formations dispensées. Je pense, notamment, à la mesure prévoyant qu'un organisme titulaire d'un agrément ne puisse sous-traiter l'exécution des prestations de formations à destination des élus financés par le DIFE qu'à la condition de justifier la nécessité de cette sous-traitance, comme le besoin d'un savoir particulier ou d'une expertise. Je veux aussi mentionner l'interdiction de la sous-traitance de second rang des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux, afin d'éviter un contournement des exigences de qualité. Enfin, je rejoins la position de la commission lorsque celle-ci a souhaité garantir la stabilité du système de formation des élus, notamment en stipulant que le Conseil national de la formation des élus locaux doit privilégier, dans les propositions de retour à l'équilibre qu'il formule au ministre chargé des collectivités territoriales, les leviers qui sont le moins attentatoires aux droits acquis des élus.

nous voici devant un problème simple à énoncer, mais complexe à résoudre : nous souhaitons mieux et davantage former les élus, mais les moyens disponibles sont trop faibles et mal utilisés. Ce projet de loi de ratification vise à gommer quelques anomalies et à améliorer certains fonctionnements, mais sans avancer suffisamment dans la réforme de la formation des élus.

Le premier, instauré en 1992 et financé par les collectivités à hauteur d'un plancher de 2 % des indemnités perçues par les élus, permet le financement de formations liées à l'exercice du mandat. Ce système est largement sous-utilisé, près de deux tiers des collectivités territoriales ne dépensant pas ces crédits budgétés, ou ne les dispositif, datant de 2015, a instauré un réel droit individuel à la formation des élus locaux, à hauteur de 1 % des indemnités perçues. Destiné initialement principalement à financer des formations liées à la reconversion des élus, il permet des formations en lien, ou pas, ou pas, avec l'exercice du mandat, et cumulables sur cinq ans. Les abus des structures de formation sont connus et dénoncés. Celles-ci réalisent une véritable captation du marché de la formation des élus : ainsi, deux organismes ont capté, en 2019, quelque 40 % du financement du DIFE. Il y avait donc urgence à réguler le marché des formations. J'insiste sur le caractère réel de l'accès à la formation et son égal accès : il existe des inégalités de formation en fonction des territoires, de la taille des communes, mais aussi parfois entre les élus majoritaires et minoritaires. J'insiste aussi sur la visibilité limitée du montant annuel des droits de formation pour chaque élu, en raison de la méconnaissance du nombre d'élus qui auront qui auront recours à ce dispositif. À cet effet, la commission propose d'instaurer une visibilité à trois ans de ces montants dès 2023, ce qui est souhaitable. La formation est un élément majeur pour l'exercice du mandat de l'élu, mais elle manque de financement. La diminution des coûts grâce à la rationalisation des frais de gestion élevés de la Caisse des dépôts et consignations Les montants et cumuls envisagés, aujourd'hui insuffisants, détournent clairement le DIFE de l'une de ses fonctions initiales primordiales : aider à la reconversion des élus en fin de mandat. Pour cela, nous demandons et attendons depuis longtemps une vraie loi et un vrai projet sur le statut de l'élu. Faute d'un contrôle suffisant, le recours généralisé à la sous-traitance a pu priver d'effet bénéfique l'agrément demandé et accordé aux organismes de formation. Le texte vise à imposer de nouvelles obligations et une certification de qualité aux organismes concernés, pour mettre fin aux dérives nuisant à la qualité des formations. Si les abus sont évidemment à combattre dans la facturation des formations, il convient de s'assurer que les droits des élus permettront un accès réel à ces dernières.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, on dénombre sur notre territoire quelque 500 000 élus locaux. Pour faire face à la complexité et à la technicité croissantes des compétences que requiert l'exercice de leur mandat, mais aussi pour préparer leur retour à une vie professionnelle, la loi a établi deux dispositifs de formation. Le premier, introduit par la loi du 3 février 1992, dont notre collègue, Jean-Pierre Sueur, alors secrétaire d'État chargé des collectivités locales, est l'auteur, prévoit que les collectivités doivent budgéter chaque année un montant minimum équivalant à 2 % des indemnités dues aux élus, dans le but de financer des formations pour eux en lien avec l'exercice de leur mandat. Le second, plus récent puisqu'il date de 2015, là encore créé par notre collègue Sueur et vous-même, madame la ministre, instaure un droit individuel à la formation des élus, le DIFE, abondé par les indemnités des élus locaux à hauteur de 1 % et géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il ouvre plus largement droit à des formations non seulement en lien avec le mandat, mais aussi avec une future reconversion professionnelle. Dans la pratique, et malgré des besoins importants pris en compte par ces dispositifs, il est apparu que ceux-ci n'ont permis qu'à une poignée d'élus de se former, que les communes les plus peuplées concentraient la quasi-totalité des efforts de formation et que le DIFE connaissait une situation déficitaire. Il était donc nécessaire de refondre le système, afin de garantir effectivement cet accès à la formation indispensable pour tous nos élus. Aussi,

Les ordonnances portant réforme de la formation des élus locaux et de ceux des communes de Nouvelle-Calédonie, que nous nous apprêtons à examiner, certes, avec un peu de retard- n'oublions pas que la crise sanitaire a quelque peu bouleversé notre agenda -, viendront faciliter et moraliser l'accès à la formation des élus locaux. faciliter, tout d'abord, grâce à la création d'une plateforme numérique permettant aux élus de mieux visualiser leurs droits et les formations auxquelles ils peuvent s'inscrire. Elles le faciliteront aussi grâce à la modification des modalités de calcul du DIFE, comptabilisé dorénavant en euros et non plus en heures, ou encore grâce à la modernisation du recouvrement du fonds du DIFE, qui se fera par un prélèvement à la source des cotisations des élus. en renforçant les prérogatives du Conseil national de la formation des élus locaux et de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion du fonds du DIFE, et le maintien de son équilibre financier, ou encore en instaurant un contrôle plus accru des organismes de formations aptes à délivrer les formations aux élus locaux, afin d'éviter les abus. Nous nous félicitons de ce que la commission- je souligne la qualité du travail de Mme la rapporteure -ait adopté l'amendement de notre collègue Alain Richard visant à anticiper les problèmes qui auraient pu se poser au moment de la transition. Cet amendement tend à prévoir que les formations entamées avant le 22 juillet 2021 puissent se dérouler jusqu'à la fin de l'année. L'adoption d'une telle mesure assurera, à n'en point une sortie plus douce du système actuel, tant pour les élus titulaires de droits que pour les organismes de formation. Je tiens enfin à rappeler ici l'importance de la formation des élus dans les collectivités d'outre-mer, de par leur éloignement géographique, sont, au même titre que les territoires ruraux, confrontés à une ingénierie souvent plus modeste, à des difficultés réelles lorsque la collectivité est récente- je pense, bien évidemment, à mon territoire, Mayotte -, ou encore à une offre de formation moins diversifiée. Au vu de nos échanges en commission et aujourd'hui en séance, il ne fait aucun doute que ce projet de loi recueillera l'assentiment de tous. En tout état de cause, mon groupe l'adoptera volontiers.

tout au long de sa conception avec les cabinets des ministres, tout d'abord avec celui de Sébastien Lecornu, dont l'action a été déterminante, puis avec le vôtre, depuis le remaniement. Quelles raisons ont poussé le Gouvernement à réformer le système de la formation des élus locaux, sinon le constat d'un double échec ? Échec à maintenir les coûts de formation à un niveau raisonnable, avec quelques organismes peu scrupuleux qui ont essoré un système ayant pu faire figure parfois de nouvel eldorado. Le rapport de l'IGA et de l'IGAS a été très explicite en la matière. Échec également de la Caisse des dépôts et consignations, qui a affiché des dépenses totalement injustifiables et disproportionnées en matière de frais de gestion du fonds de formation, auxquelles s'ajoutent des délais de réponse démesurés, voire des non-réponses. Madame la ministre, vous avez agi, et c'était nécessaire. Mais vous avez été bien plus loin que l'habilitation. Aussi, revenons-en aux termes de cette habilitation pour étudier votre réforme. Le premier point concerne l'accès au droit à la formation tout au long de la vie, le compte personnel de formation et la portabilité des droits. des droits. La fongibilité entre le DIFE et le CPF ouvre de vraies passerelles entre le parcours d'un élu et son parcours professionnel. Sur ce point, nous ne sommes pas encore parvenus à un véritable statut de l'élu, mais c'est un pas en avant qui est toujours le bienvenu. objectif de l'habilitation est de faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat. Le point central de la réforme réside dans le passage des droits ouverts en équivalent heures et non plus en euros. Je ne reviendrai pas sur le détail du calcul, mais j'insisterai sur un point de divergence que j'ai avec votre approche sur la fin du cumul du DIFE d'année en année tout au long du mandat. Tout ne se joue pas la première année, madame la ministre. J'ai donc du mal à concevoir ce qui ferait obstacle à ce cumul dans le temps. Je prends acte néanmoins de l'amendement que vous avez déposé en séance et qui me semble nature à faire l'objet d'un compromis, en introduisant un plafonnement de ce cumul. Le troisième point de l'habilitation est le référentiel de la formation et la mutualisation du financement. J'ai soulevé plusieurs interrogations quant à l'adaptabilité de ce référentiel aux problématiques nouvelles qui verront le jour et à sa nécessaire actualisation. Les réponses apportées m'ont plutôt convaincue. Nous sommes donc dans le difficile équilibre à trouver d'un côté, poser un cadre pour éviter que le contenu des formations ne dérive et, de l'autre, laisser suffisamment d'ouverture pour faire face aux besoins de formation pointue ou à l'évolutivité des matières traitées par les élus locaux. Au rang des innovations intéressantes se trouve l'abondement du compte des élus par leurs collectivités, ce qui permet à la collectivité d'honorer son obligation de formation hors DIFE, mais aussi la possible intercommunalisation. En cela, je crois que le Gouvernement répond de façon opérationnelle à nos exigences. quatrième et dernier axe de la réforme est d'assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation, ainsi que de renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation. Ce point suscite davantage d'interrogations.

Pour finir, j'y insiste, la Caisse des dépôts et consignations devra rendre des comptes sur sa gestion. C'est un point dur sur lequel nous ne devons pas céder, chers collègues, compte tenu des leçons du passé. De plus, j'ai noté l'engagement du Gouvernement sur un délai de réponse de sept jours à propos des dossiers de demande de prise en charge, ce qui est osé dans un contexte où la dématérialisation des procédures ne réglera pas tout, puisqu'un certain nombre d'élus locaux ne sont pas outillés ou connectés. Mes chers collègues, le groupe du RDSE votera en faveur de cette réforme si nous parvenons aujourd'hui à un compromis. La parole

Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la ratification de ces ordonnances, dont les objectifs initialement fixés étaient assez ambitieux. Le résultat du travail à huis clos du Gouvernement, méthode que nous ne cessons de dénoncer, est néanmoins décevant et risque fort de laisser les élus sur leur faim. Face aux dysfonctionnements des dispositifs de formation actuels, des réponses fortes étaient attendues. Si nous approuvons plusieurs mesures, nous estimons qu'elles sont insuffisantes, voire qu'elles participent à la confusion. Le travail en commission, grâce à l'adoption, notamment, de certains de nos amendements, a amélioré le texte en préservant des garanties quant aux droits des élus, comme leur cumulabilité, en donnant à ces derniers une meilleure visibilité, en offrant ou encore en renforçant les obligations des organismes de formations ajoutées par les ordonnances. Cela étant, rendre possible des abondements de la part des collectivités ou des élus eux-mêmes pour renflouer le gouffre financier du fonds pour le droit individuel à la formation des élus ne freine pas les inquiétudes. Comment des communes qui ne respectent déjà pas leur obligation légale de financer la formation de leurs élus pourraient-elles, en plus, financer le DIFE ? Cela ouvre la voie aux inégalités entre les collectivités qui en seront capables et celles qui ne le pourront pas, donc aux inégalités entre élus.

La gestion en euros, et non plus en heures, permettra de limiter les abus des organismes. Mais les élus craignent que les nouvelles règles aient un impact négatif sur leurs droits et sur le montant de leur cotisation. La rémunération que s'accorde la Caisse des dépôts et consignations pour gérer le DIFE à hauteur de 25 % de l'enveloppe du fonds sera-t-elle revue à la baisse malgré la création de la plateforme numérique ? Si les ordonnances ne suscitent pas d'avis défavorable, elles soulèvent des interrogations. Depuis la loi de 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les compétences des collectivités ont gagné en technicité. C'est pourquoi nous souhaitons réaffirmer le droit à la formation des élus créé par cette loi et nous déplorons que le financement de ce dispositif par les collectivités, qui sont tenues par la loi d'y consacrer entre 2 % et 20 % des indemnités des élus, soit sous-exécuté. Le non-respect de cette obligation touche inégalement les collectivités. Les communes sont principalement concernées, et plus d'une sur deux n'a engagé aucune dépense de formation en 2018. Mais celles de plus de 200 000 habitants y consacrent 1,9 % des indemnités, contre 0,4 dans celles de moins de 500 habitants. Le coût de la formation pour ces petites communes peut se révéler prohibitif. Très souvent, les élus ne souhaitent pas faire passer leur propre formation avant des priorités d'intérêt général.

Cette problématique étant ignorée par le texte, nous avons proposé de réparer cet oubli. En 2015, nous avons créé un second dispositif, le DIFE, financé par une cotisation obligatoire de 1 % des indemnités des élus. Cette voie indépendante de la collectivité permet aux élus de recevoir également des formations sans lien avec leur fonction, donc de favoriser leur réinsertion professionnelle. Ces deux dispositifs se complètent et sont nécessaires pour démocratiser la fonction d'élu. Sa complexité croissante peut freiner les citoyens à s'engager, d'où la nécessité que les élus soient formés afin de ne pas réserver l'élection aux « élites » et aux technocrates. Parallèlement, la réinsertion professionnelle anticipe l'après-mandat et doit permettre un brassage des représentants politiques. Nous constatons un déséquilibre entre les deux types de formations permises par ces dispositifs : celles qui sont liées à la reconversion professionnelle sont très peu utilisées et ne représentent que 3 % des demandes au titre du DIFE. Cette tendance est dommageable pour les élus et pour la démocratie. En l'état, le texte n'est pas selon nous à la hauteur de ses ambitions. Il aurait mérité un travail incluant davantage le Parlement. Notre groupe préférera donc s'abstenir.

sur les conditions d'exercice des mandats locaux, j'étais loin d'imaginer que, au siècle suivant et quelques décennies plus tard, je continuerai à parler du même sujet Cette loi fut fondatrice : auparavant, il n'y avait pas de droit à la formation pour les élus locaux, non plus d'ailleurs que de droit à la retraite.

Je crois que nous avons bien fait de créer ce droit individuel à la formation. Néanmoins, le réalisme doit nous inciter maintenant à reconnaître que, si le principe est bon,

le dispositif doit désormais être beaucoup mieux encadré, pour des motifs financiers évidents et en raison de dérives que nous avons pu constater et qui ont été déjà soulignées. Cette proposition de loi, madame la ministre, est donc nécessaire, et nous y souscrirons pour l'essentiel, comme nous le manifesterons par notre vote. J'insisterai, et mon collègue Éric Kerrouche y reviendra également, sur la question de l'agrément des organismes. des organismes. En 1992, je n'étais pas partisan que les partis politiques puissent créer des instances de formation. J'étais minoritaire, y compris au sein du Gouvernement, on peut le dire maintenant. Je suis donc attentif au fait que, cela étant désormais possible,

Pour ce qui est du DIFE, 50 % de la dépense est affectée à la formation de 14 % des bénéficiaires.

Ce pragmatisme, c'est le recours à l'intercommunalité. Veuillez conclure, mon cher collègue. Je conclus, monsieur le président, vous le voyez bien ! En l'état actuel des choses, on ne peut pas demander davantage aux communes. En revanche, la mutualisation

qui vous a invitée à mieux cadrer les dispositions d'agrément. Il a même eu la courtoisie de nous faire part des réflexions ou des interrogations

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chacun sait que la formation est un enjeu essentiel, tant pour les élus que pour les agents territoriaux. Je me réjouis donc que le présent projet de loi vienne ratifier deux ordonnances et apporte une réponse aux difficultés d'un dispositif considéré par beaucoup comme largement insatisfaisant.

sur le terrain, moins de 3 % des élus locaux suivent annuellement une formation, et les collectivités n'y consacrent en moyenne que la moitié des sommes que la loi les obligerait à budgéter. En outre, si le texte de 2015 a permis un octroi des heures dès le début du mandat, il limitait cependant la prise en charge des frais. J'ajoute que la réforme de la formation des élus est devenue particulièrement opportune avec l'arrivée de la crise sanitaire, compte tenu des défis que la situation impose aux élus. De manière l'armature financière globale du système de formation souffre de nombreux dysfonctionnements Le premier de ces dysfonctionnements se caractérise par une contradiction inhérente entre la réalité de cette organisation financière et la volonté partagée de l'exécutif et du législateur de renforcer l'accès à la formation des élus. À titre d'exemple, la combinaison d'une sous-exécution chronique des dépenses potentielles, non plafonnées, du DIFE et d'une faiblesse du fonds de financement du DIFE, qui est quant à lui plafonné, entraîne une grande fragilité financière. De nombreux organismes de formation peu scrupuleux ont, par ailleurs, abusé du recours à la sous-traitance. Ces derniers n'opéraient jusqu'à présent pas de contrôle de la qualité des formations dispensées, tout en pratiquant bien souvent des tarifs exorbitants.

chargée de la gestion du fonds, dont les moyens humains demeurent par ailleurs insuffisants. Cette situation a naturellement suscité un embouteillage de dossiers, en allongeant mécaniquement l'ensemble des délais. Ces difficultés, et bien d'autres, justifient une réforme dont les ordonnances aujourd'hui proposées à la ratification constituent le cadre. Face aux défaillances constatées du système, les objectifs définis premier de ces objectifs visait, entre autres, à « permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue » à celui qui existe en droit commun. Le deuxième était de faciliter l'accès des élus locaux à la formation. Le troisième prévoyait de « définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires »- on sait ce qu'il en est des inégalités à cet égard -et de « mutualiser le financement entre les collectivités Le dernier objectif était d'« assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux

en vue de renforcer les garanties relatives aux droits des élus à la formation ; d'améliorer la prévisibilité financière du système ; d'affermir le contrôle des organismes de formation et même parfois les rendre effectifs,

de l'élu. Le satisfecit ne saurait être complet. En effet, la réforme a une connotation trop budgétaire. Elle excède pour partie le champ de l'habilitation accordée au Gouvernement par le Parlement. Elle s'inscrit dans la perspective d'un statut de l'élu qui n'existe qu'en creux.

deux critères permettent de marquer la professionnalisation : tout d'abord, l'exercice d'une activité rémunérée ; ensuite, une formation spécifique pour remplir cette activité. L'actuel statut de l'élu fait comme si cette formation ne participait pas de la professionnalisation. Il faut rompre avec cette logique et construire, enfin, un statut de l'élu qui permette une

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les ordonnances dont ce projet de loi nous propose la ratification étaient largement attendues par les élus locaux. Elles visent juste lorsqu'elles opèrent, à la fois,

la commission des lois a fait le choix d'accepter cette ratification. À titre personnel, j'approuve naturellement cette position. En effet, dès lors que seule une très faible minorité d'élus locaux recourt actuellement au DIFE et que, par ailleurs, le budget

seront comptabilisés non plus en heures, mais en euros, afin d'induire une diminution du prix moyen des heures de formation dispensées. C'est également ce qui est prévu lorsque sont introduites de nouvelles modalités de cofinancement des formations des élus locaux, que ce soit par les collectivités locales, qui pourront abonder le compte DIFE après délibération, ou par les élus eux-mêmes, qui pourront abonder leur compte DIFE de droits issus de leur compte personnel de formation.

aussi la possibilité pour la CDC de consentir, en cas de déséquilibre du fonds DIFE, une avance de trésorerie. Dès lors, on peut assurément envisager avec confiance une meilleure réponse, à l'avenir, à cette légitime attente des élus en matière de formation. la commission des lois a estimé que le dispositif proposé pouvait encore donner lieu à certaines améliorations. Elle a ainsi décidé, sur la proposition de Mme le rapporteur, de rétablir la possibilité de cumul du DIFE sur toute la durée du mandat des élus, afin de permettre à ceux-ci d'utiliser leurs droits sur plusieurs années. La commission a également décidé d'élargir les possibilités d'abonder le fonds à l'État, à Pôle emploi, ainsi qu'à d'autres collectivités territoriales, afin de financer au titre du DIFE des formations de réinsertion professionnelle, notamment en fin de mandat. La commission a enfin permis que les élus locaux puissent s'inscrire, dès la première année de leur mandat, à des modules de formation leur permettant d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de leur mandat. Ces modifications, madame la ministre, madame le rapporteur, sont particulièrement bienvenues et adaptées à la modification que j'ai citée : il est très important qu'un élu local en début de mandat puisse bénéficier au plus vite de la formation indispensable à la mise en oeuvre de ces nouvelles attributions. Trop souvent par le passé, pour des raisons de méconnaissance ou d'indisponibilité de l'offre de formation, les élus locaux ne bénéficiaient que tardivement des formations nécessaires. Cela peut désormais être corrigé. De même, à l'approche de la fin du mandat, les élus en quête de réinsertion professionnelle pourront mieux que par le passé profiter, grâce à des financements élargis, de formations individualisées adaptées à leur profil professionnel. Cette dernière possibilité est à mon sens très importante et trouvera sa place dans dans ce statut de l'élu que nous sommes nombreux à appeler de nos voeux. Certes, la CDC doit encore mettre en oeuvre la plateforme de formation pour les élus, qui permettra un accès dématérialisé et rapide au montant de leurs droits personnels, comme aux formations éligibles.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous étudions un texte qui concerne tous les élus.

Ils siègent dans les conseils consulaires, qui sont en quelque sorte nos conseils municipaux. Répartis sur les cinq continents, ils demeurent des élus de la République attachés à l'exercice de leur mandat. La formation n'est pas seulement utile ; elle est essentielle pour nos élus locaux, d'autant que nombre d'entre eux siégeront pour la première fois en juin prochain.

mais aussi à acquérir des savoirs spécifiques, précieux dans l'exercice du mandat. Tout cela a été rappelé par les orateurs précédents. L'article 24 du décret du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires prévoit que les conseillers des Français de l'étranger reçoivent une formation pour couvrir l'ensemble de leurs domaines de compétence, avec un accès aux actions de formation organisées localement au bénéfice des personnels diplomatiques et consulaires. Pourtant, ce décret ne semble pas suffisamment appliqué depuis six ans. En effet, les élus se sont plaints régulièrement de ne pas avoir eu accès à une formation, la majorité des postes diplomatiques semblant ignorer que cette possibilité doit leur être offerte. Ce dispositif a été renforcé dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui, dans son article 111, prévoit également pour les conseillers des Français de l'étranger un droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ces formations, pilotées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, devraient être organisées à distance ou lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger. Au vu du renouvellement qui aura lieu en mai 2021, il serait bon qu'elles puissent leur être offertes au plus tard à la rentrée à la rentrée prochaine. Je voudrais également souligner la nécessité de prévoir des formations accessibles à tous, qui soient dispensées en présentiel dès que cela sera possible, afin que les conseillers puissent interagir avec leurs formateurs Cependant, j'imagine que ces élus ont aussi droit, comme tous les élus de la République, à des formations dispensées par tout autre organisme de formation agréé. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les conseillers des Français de l'étranger seraient les seuls élus à ne bénéficier que d'une seule formation, dispensée par une seule administration. Affaire à suivre, donc

Le problème de ce projet de loi est qu'il renvoie à des ordonnances dont nous ne maîtrisons pas le contenu. Comme c'est le Gouvernement qui tient la plume, il pourra en écrire et réécrire les différentes dispositions

organisent, pour le compte de leurs membres- maires, adjoints, conseillers municipaux -, des formations adaptées aux besoins qui se font ressentir sur le terrain : c'est de l'artisanat, du cousu main, du « mijoté », bref de la formation aux petits oignons, et cela pour des coûts très nettement inférieurs à ceux qui se pratiquent dans les grands cabinets.

Mon impression est que l'on veut, et c'est un peu un mal français, de nouveau tout recentraliser autour de grands cabinets ou de grandes structures, alors que, localement, on sait faire mieux et avec moins. Pour l'Association des maires du Haut-Rhin que je préside, il est tout de même plus simple de faire appel à un avocat strasbourgeois qui connaît le droit local qu'à un avocat parisien aussi « agrémenté », labellisé ou certifié qu'il soit ... Nos associations d'élus ont leurs agréments et elles sont contrôlées. Chaque élu disposait d'un quota de vingt heures de formation. Encadrer le prix de l'heure de formation est une très bonne chose, qui aurait dû être faite dès le départ, ce qui aurait peut-être permis d'éviter certains abus. Pour résumer rapidement mon propos, madame la ministre, faites confiance aux associations départementales de maires dans votre réforme de la formation des élus locaux. N'y allez ni trop vite ni trop fort

et le rôle du Conseil national de la formation des élus locaux. Nous reviendrons sur ces sujets nos amendements, mais les propositions du Gouvernement nécessitent d'être encadrées par des garanties.

élaboré au niveau réglementaire le sera de manière constructive. Sachez que je suis très sensible à votre amendement, que je considère comme un amendement d'appel,

Le Gouvernement propose dans ces ordonnances de favoriser la mutualisation du droit à la formation des conseillers municipaux au niveau des intercommunalités. Plus précisément, l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 renforce les possibilités et obligations de délibération des EPCI en matière d'exercice du droit à la formation. d'orientations communes et la mise en commun d'outils, ainsi que la participation financière à ces formations liées à l'exercice du mandat. Face aux difficultés que rencontrent de nombreuses communes pour répondre à leurs obligations en matière de droit à la formation des élus, la mutualisation peut être une solution, notamment d'un point de vue financier. Rappelons que, dans une commune de moins de 2 000 habitants, la dépense moyenne par élu n'atteint que 9 euros par an, contre 376 euros dans une commune de plus de 100 000 habitants. Nous le répétons, des solutions doivent être trouvées pour résoudre ce paradoxe inéquitable et anti-redistributif, qui dessert les petites communes. Les mairies ont déjà la possibilité de transférer à l'EPCI leur compétence en matière de formation, mais elles le font très rarement. Cette mutualisation peut permettre de rassembler les élus autour d'enjeux partagés dans une dynamique collective et de rencontre, mais les relations entre EPCI et communes et la « confiance » des élus envers ces structures risquent de freiner ce mouvement. Comme nous l'avons relevé dans le rapport sénatorial sur l'exercice des mandats locaux, les élus sont prudents et craignent une régression de leurs droits en l'absence de dispositions législatives claires sur le mode de calcul du budget « formation » en cas de mutualisation. Nous proposons donc, par cet amendement, de sécuriser juridiquement les modalités financières de mutualisation, en reprenant les règles prévues pour les communes.

est à Mme Michelle Gréaume. Le Conseil national de la formation des élus locaux, le CNFEL, est l'organe consultatif qui s'est vu confier le soin de définir les orientations des formations proposées aux élus. Cette instance régule le marché de la formation, en donnant un avis sur les décisions ministérielles d'agrément délivré aux organismes de formation. La présente ordonnance renforce le rôle du CNFEL, et les ajouts de la commission des lois le confortent également en encadrant ses nouvelles missions. devra notamment s'assurer de l'équilibre financier du fonds DIFE, formuler des propositions au Gouvernement pour le rétablir, puis donner un avis assez contraignant sur le projet de rétablissement de l'équilibre financier. Nous espérons que cette amélioration apportée par la commission demeurera dans le texte, tout comme la formulation de prévisions du montant des droits des élus. Nous tenons également au caractère public du rapport annuel qu'il devra établir sur la formation et sur la gestion du DIFE.

Nous proposons donc, par cet amendement, le rétablissement de cette précision : il nous semble important que le Conseil conserve cette parité entre personnalités qualifiées et élus. Nous en profitons également pour rappeler dans la loi que les membres du Conseil doivent représenter le pluralisme politique et l'ensemble des collectivités territoriales, afin d'y assurer au mieux la représentation de tous les élus locaux. Quel

votre commission a souhaité rétablir de manière explicite le caractère cumulable des droits accordés annuellement aux élus dans le cadre du DIFE. Je le comprends parfaitement, mais ce principe doit être concilié avec l'objectif de pérennité financière du DIFE. C'est pourquoi le Gouvernement propose que le montant global des droits cumulables puisse être plafonné, comme c'est d'ailleurs le cas pour le compte personnel de formation. Ce plafond permettra d'éviter que les droits accordés annuellement aux élus ne soient réduits par anticipation des dépenses importantes qui pourraient découler de la consommation en fin de mandat des droits accumulés. Permettez-moi d'illustrer ce qui pourrait se produire si vous ne prévoyez pas un tel plafonnement. Supposons que le nombre d'élus bénéficiaire du DIFE demeure, comme en 2020, autour de 13 000 élus et que l'enveloppe accordée annuellement aux élus s'élève à 700 euros. Au bout de six ans, la consommation des droits

abondé de différentes manières, qui sont cumulables. La collectivité peut décider d'abonder les droits de l'élu dès lors qu'elle a pris une délibération pour fixer le cadre de son intervention,

La commission a apporté des ajouts salutaires concernant la mise en place d'une prévision triennale de la valeur des droits et la primauté des propositions du CNFEL, sauvegardant la valeur des droits et la stabilité des cotisations. Mme la rapporteure porte également un amendement visant la fusion triennale des droits. Cette disposition est tout à fait salutaire.

des formations sont organisées par les associations départementales d'élus et les services de l'État, mais elles ne sont accessibles qu'aux maires. Nous proposons que, sur la plateforme,

nécessitant de recourir à une expertise très pointue, pour un temps limité, qui n'existerait pas dans un organisme de formation. Par exemple, les élus suivent une formation à l'urbanisme,